Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour un rappel au règlement.

sur les ventes d'armes au régime criminel d'Arabie saoudite. Non seulement le régime d'Arabie saoudite et le dauphin de l'émir dictateur qui commande dans ce pays de l'émir dictateur qui commande dans ce pays sont à l'origine d'un crime absolument odieux, digne du Moyen Âge, mais de surcroît les dirigeants de ce pays commettent de multiples crimes de guerre contre les Houthis au Yémen.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi a pour objet de répondre à une revendication de longue date des associations de soutien aux personnes handicapées.

C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité reprendre la proposition de loi déposée par Marie-George Buffet à l'Assemblée nationale le 6 décembre 2017 et cosignée par une cinquantaine de députés de toutes sensibilités politiques. Visiblement, la situation a évolué, « régressé » serait le mot juste, puisque notre proposition de loi n'a pas été votée en commission par les autres groupes, à l'exception du groupe socialiste. Pourtant, cette proposition de loi est plus que jamais d'actualité. Elle permettrait non seulement d'octroyer aux personnes handicapées un complément de revenu, mais également de compenser, autant que faire se peut, les difficultés financières liées au handicap. Nous rétablissons la mission première de l'AAH, à savoir d'être une allocation de compensation. Pour rappel, plus de 1 million de personnes en France sont dans une situation de handicap telle qu'elles ne peuvent accéder durablement à l'emploi et sont, à ce titre, bénéficiaires de l'AAH. Cette allocation n'a donc pas pour objectif de fournir une aide temporaire, comme les minima sociaux tels que le RSA, afin d'empêcher la situation de la personne de trop se dégrader. Il s'agit bien, ici, d'une ressource financière permettant de pallier une situation qui n'a que peu de chances, hélas ! d'évoluer dans un sens meilleur. C'est d'ailleurs ce que montrent les statistiques, puisque 90 % des allocataires renouvellent leur demande d'AAH. Autrement dit, pour la quasi-totalité des bénéficiaires de l'allocation, il n'y a pas de perspective d'amélioration de leur état de santé. L'AAH est donc bien un droit, une allocation visant à protéger celles et ceux qui sont placés en situation de vulnérabilité et à compenser les difficultés rencontrées au quotidien. La vulnérabilité à laquelle sont confrontées les personnes en situation de handicap est bien réelle. Ainsi, un article de l'Observatoire des inégalités, publié en octobre 2017, rapporte que la moitié des personnes dont le handicap est reconnu administrativement ont un niveau de vie mensuel inférieur de quasiment 200 euros à celui des personnes n'ayant pas de handicap. Plus le handicap est sévère, plus l'écart se creuse, allant jusqu'à 500 euros. Les deux revalorisations de l'AAH annoncées par le Gouvernement ne permettront pas de supprimer cet écart ni de porter l'AAH au niveau du seuil de pauvreté, fixé à 1 026 euros- faut-il le rappeler ? Cette exposition plus forte des personnes en situation de handicap à la pauvreté et à la précarité n'est malheureusement pas près de diminuer. En effet, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui précarisent davantage celles et ceux qui sont déjà en situation de grande fragilité. J'en citerai quelques-unes : suppression du complément de ressources ; baisse du quota d'appartements adaptés, c'est-à-dire accessibles, dans les constructions neuves ; limitation du cumul entre RSA et AAH AAH ; suppression de l'aide au transport pour les enfants et adultes handicapés. Et cette liste est loin d'être exhaustive ! À ces mesures, profondément injustes, s'ajoutent celles qui concernent tout un chacun : la baisse des APL, la hausse de la CSG ou encore la désindexation de nombreuses prestations sociales. Aussi est-il urgent d'agir maintenant, non seulement afin d'améliorer le niveau de vie des personnes en situation de handicap, mais également pour une question de droits fondamentaux. L'AAH est une allocation d'autonomie qui, bien qu'insuffisante, a pour but de donner à son bénéficiaire les moyens de son indépendance financière. Prendre en compte les revenus du conjoint ou de la conjointe a des conséquences extrêmement fâcheuses. Certains des bénéficiaires, en effet, voient leur allocation tellement diminuée qu'elle ne leur permet pas de vivre décemment. D'autres en sont tout simplement privés ! Leur subsistance et leur qualité de vie dépendent donc entièrement de leur conjointe ou de leur conjoint, ce qui les place dans une situation de dépendance pouvant s'avérer humiliante. C'est d'ailleurs le phénomène qui est décrit dans un reportage du journal télévisé de France 3 diffusé en mars dernier. On y voit un homme expliquer que, depuis son mariage, l'AAH qu'il percevait a été supprimée, ce qui ne lui laisse pour subsister qu'une pension d'invalidité de 330 euros. Cette situation l'oblige à « vivre aux crochets de sa femme », il ne peut faire aucun projet, il ne peut pas emprunter d'argent à la banque : comme il le souligne lui-même, « en tant que personne », il ne peut rien faire. Dans ce reportage, il s'agit d'un homme, mais la problématique de la dépendance au conjoint ou à la conjointe se pose de manière encore plus grave pour les femmes handicapées. En France, le nombre de femmes handicapées est quasiment aussi élevé que le nombre d'hommes. Pourtant, les femmes font bien moins souvent l'objet d'une reconnaissance administrative de leur situation, puisqu'elles ne constituent que 40 % des bénéficiaires de l'AAH. Par ailleurs, selon une étude menée par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, publiée le 16 mars 2016, les femmes handicapées sont celles qui sont le plus victimes de violences physiques et sexuelles au sein du couple. Pour ces femmes, l'arrêt de la prise en compte du revenu du conjoint dans l'AAH est une nécessité afin qu'elles puissent retrouver leur indépendance et s'émanciper de situations parfois destructrices. destructrices. C'est pourquoi notre proposition de loi est soutenue non seulement par les associations d'aide aux personnes en situation de handicap, mais aussi par les associations féministes. Je pense tout particulièrement à l'association Femmes pour le dire, femmes pour agir, fondée par Maudy Piot, militante inlassable des femmes handicapées, féministe reconnue, décédée, hélas ! le 25 décembre dernier. Elle se battait pour que les femmes handicapées jouissent de leurs droits de citoyennes, ce qui est le sens même de notre proposition de loi. Il est fondamental de bien comprendre que l'AAH est une allocation attachée à la personne et qu'elle ne saurait être retirée en cas de vie de couple. La pension d'un retraité ne dépend pas des ressources de son conjoint que je sache ! Je défends par ailleurs avec les associations féministes l'individualisation des droits sociaux garantissant une indépendance économique des femmes.

Le texte aujourd'hui soumis à votre examen a fait l'objet en commission des affaires sociales d'un débat nourri et utile, à l'issue duquel un problème demeurait entier : quelle est la nature de l'allocation aux adultes handicapés ? Cette allocation occupe une place à part dans le paysage des prestations sociales attribuées aux personnes handicapées. Elle est versée aux personnes handicapées dont l'incapacité permanente les tient durablement éloignées de l'emploi. Depuis sa création par la loi fondatrice du 30 juin 1975, l'AAH a toujours été perçue comme un minimum social, autrement dit comme un revenu de remplacement versé par les pouvoirs publics aux personnes bénéficiaires en vertu de la solidarité nationale, en subsidiarité des autres formes de solidarité. C'est la raison pour laquelle les modalités d'attribution de l'AAH présentent une certaine parenté avec celles du revenu de solidarité active. Il s'agit, en effet, d'une prestation sociale différentielle, qui part non pas du besoin de la personne qu'elle finance, mais d'un revenu minimum qu'elle lui garantit. Elle tient compte des revenus du conjoint, suggérant ainsi que l'accompagnement d'une personne handicapée durablement écartée du marché du travail serait moins coûteux lorsque cette dernière est en couple que lorsqu'elle vit seule. Ces caractères de l'AAH sont bien connus et traduisent l'esprit d'une époque où l'accompagnement du handicap s'entendait comme le prolongement d'une forme de charité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis une autre grande loi, celle du 11 février 2005, une autre logique d'intervention publique auprès des personnes handicapées s'est affirmée : la logique de compensation. Contrairement à la logique de solidarité, la compensation ne vise pas à assurer à la personne handicapée un revenu de remplacement dans le but de maintenir son niveau au-dessus d'un certain seuil, objet de financer, sans considération de ressources ou de foyer, l'indemnisation du « préjudice moral » que subit la personne dans ses difficultés quotidiennes du fait de son handicap. Cette indemnisation est en grande partie assurée par la prestation de compensation du handicap, attribuée par les conseils départementaux. Le financement de l'accompagnement de la personne handicapée se situe au croisement de ces deux philosophies, solidarité et compensation, ce qui peut parfois en rendre la compréhension malaisée. Individuel et déconnecté du niveau de revenu lorsqu'il s'agit de compenser le besoin en aides humaines et techniques consécutif à un handicap, le financement prend des formes plus solidaristes, proches de la logique des minima sociaux,

Au nom de quoi un handicap ferait-il appel au devoir d'indemnisation des pouvoirs publics, dans certains cas, et à l'obligation solidaire d'un minimum social, dans d'autres ? De toute évidence, pour des motifs liés autant à son histoire qu'aux tâtonnements récents des politiques publiques en matière de handicap, nous peinons encore à faire un choix clair. La commission des affaires sociales du Sénat a longuement débattu sans parvenir à trancher. Même nos collègues défavorables à la proposition de loi ont bien été contraints de reconnaître qu'une pareille dualité, en plus de plonger dans la confusion certains de nos concitoyens les plus fragiles, était le signe d'une politique publique inaboutie et vacillant sur ses propres principes. Ce texte tend à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul et dans l'attribution de l'AAH afin afin de la faire résolument entrer dans la catégorie des prestations de compensation. On dit de ce texte qu'il dénature profondément l'AAH. Mes chers collègues, c'est tout le contraire ! Nous mettons simplement nos pas dans ceux du législateur de 2005, qui a posé le principe compensateur comme référence unanimement acquise aujourd'hui. Au même titre qu'une aide humaine ou une aide technique compense la perte d'autonomie liée au handicap, nous estimons logiquement que l'AAH compense la perte de revenu liée à l'incapacité de s'insérer durablement sur le marché du travail. Son attribution doit donc obéir à des principes de compensation. Pourquoi voir une aberration là où il n'y a que bon sens et désir de simplifier la vie de personnes qui n'ont vraiment pas besoin de complications ? Notre texte est donc utile, mais il est aussi indispensable, surtout en cette période où s'ouvre la discussion budgétaire. Le projet de loi de finances de l'an dernier avait effectivement permis au Gouvernement de faire l'annonce de deux mesures relatives à l'AAH, dont l'une ne laisse pas de nous inquiéter. La première mesure concerne la revalorisation du montant individuel maximal auquel un bénéficiaire peut prétendre. De 820 euros actuellement, ce plafond passerait progressivement à 900 euros en novembre 2019, ce dont nous nous félicitons. En revanche, la seconde mesure prévoit l'abaissement du plafond de ressources en deçà duquel un bénéficiaire en couple peut toucher l'AAH. Ce plafond, qui est actuellement le double du plafond individuel, va se voir appliquer un coefficient dégressif, illustrant ainsi l'ambition du Gouvernement de « familialiser » une prestation qui doit à tout prix rester individuelle. Nous avons, à maintes reprises, questionné la direction générale de la cohésion sociale sur les impacts chiffrés de ces deux mesures, jamais reçu de réponse. Or nous avons toutes les raisons de craindre que, malgré la bonne nouvelle de la revalorisation, l'abaissement du plafond ne manquera pas d'exclure certains allocataires d'un dispositif dont ils bénéficient actuellement. Nous en avons en tout cas la preuve irréfutable par les chiffres pour le cas d'un couple composé de deux bénéficiaires de l'AAH. Mes chers collègues, c'est tout le contraire de l'ambition de notre texte. Il ne s'agit pas ici d'une mesure que l'on pourrait accuser d'être naïvement généreuse, il s'agit d'un pas nouveau franchi vers une politique publique du handicap plus cohérente, plus lisible et plus juste. La parole

Madame la présidente, madame la sénatrice Laurence Cohen, madame la rapporteur, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de me donner, par cette proposition l'occasion de partager une nouvelle fois avec vous l'engagement total du Gouvernement en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Cette priorité du quinquennat sera de nouveau mise à l'honneur lors du comité interministériel du handicap que réunit le Premier ministre demain matin, à Matignon. J'espère que vous me donnerez l'occasion de vous présenter les mesures importantes qui en seront issues, par exemple lors d'une prochaine séance de questions d'actualité. Je veux d'abord rappeler que cette priorité se traduit très concrètement par un effort financier sans précédent

Quel est le sens de cette revalorisation et comment s'articule-t-elle avec l'ensemble de la politique du handicap du Gouvernement et avec notre projet de société inclusive ? C'est une question centrale pour l'examen de votre proposition de loi, madame la sénatrice Cohen, que je voudrai éclairer par mon propos. Depuis sa création, en 1975, l'allocation aux adultes handicapés est un minimum social. Elle vise à assurer un minimum de ressources aux personnes auxquelles leur handicap interdit de travailler Elle n'a, en conséquence, aucune vocation à « compenser » le handicap, d'autant qu'une prestation a été spécifiquement créée à cette fin depuis 2005 : la prestation de compensation du handicap sur laquelle L'AAH, en qualité de minimum social, est la manifestation de la solidarité nationale envers les plus démunis, ce qui justifie pleinement qu'elle soit financée par le budget de l'État. Avec le RSA et l'ensemble des autres prestations sociales, l'AAH participe pleinement de notre « filet de sécurité » et contribue fortement à la réduction de la pauvreté monétaire dans notre pays. Il faut s'en féliciter, c'est un filet solide Les transferts sociaux et fiscaux diminuent le taux de pauvreté en France de 8 points ; les seuls minima réduisent l'intensité de la pauvreté de plus de 6 points. aussi le rappeler, c'est un filet compliqué- comme vous l'avez parfaitement souligné, madame la sénatrice -, dont la complexité même peut s'opposer à l'accès aux droits des personnes. C'est la raison pour laquelle, je veux le rappeler, le Gouvernement s'est engagé, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, que pilote Agnès Buzyn, à mener un chantier de refonte des minima sociaux dans la perspective de la mise en place d'un revenu universel d'activité. Ce chantier et cette vision d'ensemble sont en effet indispensables pour rendre plus équitable et plus incitatif à l'activité un système aujourd'hui complexifié par la coexistence de dix minima. Une grande concertation nationale et citoyenne sera organisée en ce sens de janvier à juin 2019. Mais puisque votre proposition, madame la sénatrice, se concentre sur la seule allocation aux adultes handicapés, arrêtons-nous sur elle. Oui, cette prestation s'articule avec les solidarités familiales, notamment la solidarité entre époux reconnue par le droit civil, car c'est un principe de base de notre modèle social. Ainsi, comme tous les minima sociaux, l'AAH est assortie d'une condition de ressources. Si le bénéficiaire dispose de ressources personnelles ou s'il peut compter sur le soutien financier des autres membres de son foyer au titre de la solidarité familiale, la priorité doit être donnée à la mobilisation préalable de ces ressources. C'est à ce titre que les ressources du conjoint sont prises en compte dans le calcul de l'AAH. Vous le comprenez, mesdames, messieurs les sénateurs, revenir sur cette articulation des solidarités, supprimer la condition de ressource appréciée à l'échelle du foyer, comme le prévoit la proposition de loi de Mme la sénatrice Cohen, reviendrait donc sur la nature même de l'allocation aux adultes handicapés. aux adultes handicapés. Ne nous y trompons pas : la prise en compte de la composition du foyer du bénéficiaire dans le calcul de la prestation s'exerce bien au bénéfice des personnes dès lors que le plafond de ressources pour bénéficier de l'AAH augmente, parallèlement à la taille du foyer. cela veut dire que le plafond de ressources est plus élevé lorsque le bénéficiaire est en couple, comme il l'est lorsque le bénéficiaire a des enfants. Ainsi, un bénéficiaire de l'AAH en couple, sans revenu d'activité propre, peut continuer de percevoir cette allocation jusqu'à ce que les ressources de son conjoint atteignent 2 169 euros mensuels, soit 1,8 SMIC. 1,8 SMIC. Dans le cas où c'est l'allocataire de l'AAH qui travaille, et pas son conjoint, les règles actuelles de « conjugalisation » permettent à ce bénéficiaire de cumuler son allocation à taux plein en complément, par exemple, d'un SMIC. En novembre 2019, cet allocataire pourra percevoir 900 euros en complément de son revenu d'activité au SMIC. Si l'on ne prend plus en compte les ressources à l'échelle du foyer, cet allocataire ne pourra plus prétendre qu'à 344 euros mensuels. C'est un manque à gagner très important de 556 euros par mois pour ce foyer. Si je salue bien volontiers le travail et la volonté de Mme la sénatrice Laurence Cohen dans l'élaboration de ce texte, je me dois d'alerter sur les conséquences de sa proposition. En supprimant le plafond de ressources pour les couples, elle aurait pour première conséquence de diminuer le montant de l'allocation de certains bénéficiaires de l'AAH en couple, puisque ne serait plus retenu que le plafond pour les personnes seules. Ainsi, paradoxalement, cette mesure, dont l'impact budgétaire est évalué à près de 360 millions d'euros par an, ferait certes des gagnants, mais aussi 57 000 ménages perdants, avec des gains et pertes mensuelles très importants. Vous le savez aussi, mais il n'est pas inutile de le rappeler, les modalités de calcul de l'AAH prennent pleinement en compte les besoins spécifiques de ses bénéficiaires. Tout d'abord, une « base ressources » réduite : le calcul du droit à l'AAH ne prend en compte que les seules ressources soumises à l'impôt sur le revenu. un mécanisme d'intéressement à la reprise d'une activité particulièrement incitatif : les allocataires bénéficient d'un cumul intégral de leurs revenus avec l'AAH pendant les six premiers mois de la reprise d'un emploi ; ils peuvent ensuite cumuler revenus d'activité et AAH selon un mécanisme d'abattement avantageux. un abattement spécifique de 20 % est prévu pour la prise en compte des revenus du conjoint. Cela signifie concrètement que, si vous êtes bénéficiaire de l'AAH et que votre conjoint gagne 1 500 euros mensuels, seuls 1 200 euros sont pris en compte pour le calcul de vos droits. Enfin, le plafond de ressources prévu est supérieur à celui applicable à d'autres minima sociaux. D'autres dispositifs et droits connexes supplémentaires viennent également répondre à la spécificité des besoins des personnes en situation de handicap. des exonérations fiscales spécifiques sont prévues en matière de taxe d'habitation et de taxe foncière, sous condition de ressources et de cohabitation. Les bénéficiaires de l'AAH bénéficient également d'une aide à une complémentaire santé que la ministre des solidarités et de la santé revoit et améliore substantiellement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, conformément aux annonces de la stratégie de lutte contre la pauvreté. L'ensemble de ces règles et de ces droits connexes ont été conçus pour soutenir l'autonomie des personnes. Cet objectif reste pleinement celui du Gouvernement, comme l'illustre l'investissement social massif que nous faisons en direction des bénéficiaires de l'AAH. Afin de lutter contre la pauvreté subie des personnes en situation de handicap, le projet de budget pour 2019 sera marqué, pour la deuxième année consécutive, par la revalorisation exceptionnelle de l'allocation, conformément à l'engagement du Président de la République. Il s'agit d'une hausse sans précédent, dont vous connaissez les modalités. Elle représente un investissement de plus de 2 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat. Cela représente une hausse totale de l'AAH de 11 % par rapport à son montant actuel. C'est l'équivalent d'un treizième mois pour les personnes concernées, qui sont- je veux le rappeler -plus de 1 million, l'AAH représentant le deuxième minimum social par le nombre de ses bénéficiaires. Cette hausse répond à l'engagement du Président de la République de renforcer la solidarité nationale en direction de ceux qui en ont le plus besoin. Mais il ne s'agit pas de compenser le handicap, comme je l'indiquais en introduction, car cette compensation relève non pas de l'AAH, mais davantage de la prestation de compensation du handicap, introduite en 2006. La PCH est une prestation en nature visant à contribuer au financement des besoins de compensation, à domicile et en établissement, en complément des aides de la sécurité sociale. Il s'agit d'une prestation personnalisée, fondée sur une évaluation multidimensionnelle des besoins de chaque personne et prenant en compte son projet de vie. Il s'agit d'une prestation universelle, quasiment sans condition de ressources, attribuée par les maisons départementales des personnes handicapées et financée par les départements, avec le concours de la solidarité nationale.

La refonte de la prestation doit notamment mieux soutenir la parentalité des personnes en situation de handicap. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons évoqué des prestations, des dispositifs, des règles techniques et des chiffres, mais il me semble important de conclure en rappelant au-delà d'un accès simplifié et plus équitable à ces prestations et compensations, le soutien à l'autonomie des personnes handicapées et à leur pleine participation à la société et à la citoyenneté est au coeur de la société inclusive que construit actuellement le Gouvernement, projet qui veut reconnaître dans les citoyens en situation de handicap des citoyens à part entière, et non des citoyens à part. Cette reconnaissance passe par le rétablissement de l'ensemble des personnes dans leur pleine citoyenneté, avec le plein exercice du droit de vote des majeurs protégés,

engagé en faveur de l'accessibilité universelle et sur le soutien à l'activité des personnes handicapées, confortée par les dispositions de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce projet nous rassemble largement, comme je l'ai vérifié encore récemment, lors de la présentation par le sénateur Philippe Mouiller de son excellent rapport sur le financement de la politique du handicap. Je le remercie de m'y avoir associée. C'est la raison pour laquelle, tout en émettant un avis défavorable sur cette proposition de loi, je suis confiante dans le soutien de votre assemblée pour coconstruire une société du vivre ensemble qui fasse pleinement place aux personnes et à leurs différences. La

de la très nécessaire proposition de loi portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés.

Notons que cette proposition de loi a d'abord été déposée à l'Assemblée nationale, toujours sur l'initiative des parlementaires communistes, et cosignée par de nombreux députés, issus de plusieurs groupes politiques.

nouvelle illustration, s'il en était besoin, de l'importance du Sénat dans notre vie politique et de l'importance du bicamérisme. C'est un fait dont il faudra se souvenir lors du futur examen au Parlement de la réforme constitutionnelle, qui interviendra en janvier prochain. La proposition de loi que nous examinons répond aux attentes des personnes en situation de handicap et à celles de leurs associations de défense, qui dénoncent, depuis des années, la prise en compte du revenu du conjoint. Rappelons, tout d'abord, que l'AAH bénéficiait à 1,13 million de personnes en 2017 et que, de 819 euros par mois pour une personne seule, elle atteindra 860 euros au 1 novembre 2018, puis 900 euros

revalorisation de l'AAH pour une personne seule s'accompagnera d'une baisse progressive pour les bénéficiaires en couple. Ainsi, le coefficient multiplicateur maximal est passé de 2 à 1,9 en 2018 et s'élèvera à 1,8 l'année prochaine, ce qui pourra exclure certains couples du bénéfice de l'allocation, dans des proportions dont nous ne connaissons pas l'ampleur, comme l'a regretté notre rapporteur. Les couples percevant tous deux l'AAH connaîtront eux aussi une baisse nette des revenus du foyer.

Citoyenne à part entière, la personne handicapée n'a pas demandé à être privée de sa capacité à travailler et doit, à notre sens, avoir le choix de ne pas dépendre financièrement de son conjoint. L'AAH n'est pas un minimum social comme un autre : c'est le calcul d'un degré d'invalidité, contraignant malheureusement la personne concernée à renoncer au travail. Je rappelle que, pour percevoir l'AAH, il faut se voir reconnaître un taux d'incapacité de 80 %, ce qui correspond à un handicap lourd, empêchant de travailler. Mais qui dit renoncement au travail ne dit surtout pas renoncement à une vie sociale, culturelle ou familiale ! Or, bien souvent, les personnes handicapées n'ont que l'AAH pour seule ressource. Pour mesurer les difficultés d'insertion des personnes souffrant d'un handicap, je veux insister sur un chiffre particulièrement éclairant : seuls 6 % des allocataires de l'AAH sortent du dispositif d'une année sur l'autre, d'après une étude récente. C'est dire si l'AAH, son maintien à taux plein, sa revalorisation régulière sont essentiels pour nos concitoyens touchés par le handicap. Cependant, force est de constater que le Gouvernement, au-delà des déclarations de principe et d'affichage sur la nécessité de mener une politique inclusive, n'apporte malheureusement qu'une réponse comptable, difficilement justifiable et décalée par rapport aux réalités vécues. Nous avons déjà constaté ce décalage entre l'affirmation de grands principes et la réalité concrète à l'occasion des débats parlementaires sur le projet de loi ÉLAN. En l'espèce, l'article 18 de ce texte, relatif à l'accessibilité des logements pour les personnes handicapées, prévoit que seuls 20 % des nouveaux logements collectifs leur seront accessibles, alors que la loi de 2005 prévoyait, pour ces mêmes programmes neufs, un taux de 100

Je ne demande qu'à être démentie, tout du moins aujourd'hui, madame la secrétaire d'État, en vous voyant apporter votre soutien à cette très attendue proposition de loi de nos collègues du groupe communiste républicain citoyen attendue par les intéressés, attendue par le mouvement associatif, lequel est extrêmement inquiet, attendue et espérée par nous-mêmes, sénateurs et sénatrices du groupe socialiste et républicain. L'adoption du texte ne mettrait pas en péril, tant s'en faut, l'équilibre des finances publiques- je rappelle que seuls 23 % des allocataires de l'AAH sont en couple. Ce serait un geste de solidarité, de fraternité et un bon signal envers nos concitoyens les plus exposés et les plus fragiles, déjà durement frappés par leur situation de personnes handicapées. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des sénateurs du groupe socialiste et républicain, qui ne peuvent accepter que les politiques publiques se réduisent à la recherche d'équilibres budgétaires, voteront avec détermination et enthousiasme cette proposition de loi. La parole est à Mme Véronique

nous nous réunissons aujourd'hui pour examiner une proposition qui touche à un sujet auquel nous sommes, je crois, tous sensibles : la vie quotidienne des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Attribuée à environ 1 million de personnes en situation de handicap, l'AAH prend en compte l'ensemble des ressources retenues dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Si nous sommes tous d'accord pour considérer l'AAH comme un outil indispensable à l'inclusion des personnes handicapées dans notre société, les avis divergent quant à une éventuelle réforme de son mode de calcul. Je m'efforcerai de détailler la position du groupe du RDSE sur ce sujet. Les auteurs de la proposition de loi déplorent une situation de dépendance financière des personnes handicapées à l'égard de leur conjoint, en raison du caractère dégressif de l'AAH, qui prend en compte l'ensemble des revenus du foyer. Bien sûr, nous considérons que tout doit être mis en oeuvre pour garantir le maximum d'autonomie des personnes en situation de handicap et limiter ainsi le niveau de dépendance à l'égard de leurs proches, à tous les âges de la vie. Malgré une reconnaissance croissante et heureuse de l'engagement des proches aidants- nous en discuterons demain -, c'est bien la société tout entière et dans toutes ses dimensions qui doit être aux avant-postes dans ce domaine, pour permettre l'émancipation de chacun. la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait figure de modèle et s'est imposée comme le fondement de toutes les réformes entreprises dans ce domaine. Elle pose notamment comme principes fondamentaux l'émancipation et la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap et rappelle qu'une société plus juste et apaisée est une société inclusive. La proposition de loi que nous examinons intervient dans un contexte particulier de modification des règles de l'AAH par le Gouvernement. En effet, ce dernier a annoncé plusieurs revalorisations exceptionnelles, qui porteront l'AAH à 860 euros en novembre 2018 et 900 euros en novembre 2019, ce qui équivaut à une augmentation significative de 80 euros pour les allocataires. Toutefois, nous regrettons que d'autres mesures atténuent son véritable impact. Je veux simplement évoquer la baisse du coefficient de prise en compte des revenus du conjoint, qui entraîne une baisse progressive du plafond de ressources pour les couples, ainsi que l'article 65 du projet de loi de finances pour 2019, qui propose de revenir sur l'indexation de l'AAH Nos collègues du groupe CRCE proposent de supprimer la prise en compte du revenu du conjoint dans la base de calcul de l'AAH. Nous comprenons bien la spécificité de l'AAH, laquelle permet de faire face à une situation qui, dans la majorité des cas, n'a pas vocation à s'améliorer. Toutefois, pour la plupart des minima sociaux, comme le RSA, les revenus du conjoint sont également pris en compte

Par ailleurs, selon ces mêmes auteurs, le principe de l'allocation est de garantir l'autonomie de la personne. Or l'objectif premier de l'AAH est non pas de garantir l'autonomie de son bénéficiaire, mais d'« assurer un minimum de ressources », donc de lutter contre la grande pauvreté des personnes en situation de handicap. À ce titre, il paraît cohérent, en l'état des autres prestations, de prendre en compte l'ensemble des ressources du foyer. Quant à la PCH, elle a pour objectif de compenser le handicap. Tentons de prendre un peu de hauteur sur la question : nous saluons de nouveau l'augmentation significative de l'AAH et, en même temps, nous mesurons l'ampleur du travail qui reste à accomplir. La lutte contre la pauvreté des personnes handicapées et la compensation par l'État des entraves particulières engendrées par leur situation ne sont que les parties émergées de l'iceberg. fragile et imparfait qui leur est réservé dans la société demeure un frein à leur pleine inclusion. Le handicap, aussi individuel soit-il, est accentué par la faible accessibilité des établissements recevant du public, mais aussi par la faible adaptation du marché de l'emploi et de la formation, tout comme par l'offre encore insuffisante d'activités sportives ou culturelles mises à la disposition des citoyens concernés. Dans cette vision globale, l'environnement familial et social, donc la solidarité familiale, joue bien évidemment un rôle majeur. En conséquence, penser l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap sous le seul angle de la suppression des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'AAH serait passer à côté de l'enjeu majeur des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif d'une société inclusive,

Cohen, qui tend à la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés. À titre préliminaire, je veux rappeler que cette aide financière a pour but de garantir un minimum de ressources. Elle est l'expression de la solidarité nationale.

Celle-ci s'est exprimée au Sénat au travers d'une question de notre collègue Bernard Jomier, puis a pris forme à l'Assemblée nationale, d'abord avec une première proposition de loi, déposée le 17 janvier 2018 par Laurence Trastour-Isnart, membre avec une seconde, déposée le 21 mars 2018 par Marie-George Buffet. Elle a fait d'ailleurs l'objet d'une adhésion transpartisane. Le texte a été renvoyé en commission des affaires sociales, et non en commission spéciale, contrairement à ce qu'avait souhaité le groupe Gauche démocrate et républicaine. Je prends note de l'opposition formée par la présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, et je la regrette. En effet, j'estime qu'il eût été préférable d'aboutir à la constitution d'une telle commission. Celle-ci aurait permis à la représentation nationale d'envoyer un message politique clair à destination de nos concitoyens

De plus, elle aurait permis de mener une réflexion pluridisciplinaire, d'avoir une vision globale sur l'application de cette proposition et, probablement, d'envisager une réforme de plus grande ampleur sur le sujet. J'y reviendrai dans quelques instants. En ce qui concerne nos débats, je veux avant tout saluer les travaux de notre collègue rapporteur. Nous rejoignons le constat qu'elle a dressé et sa présentation de la philosophie dans laquelle s'inscrit cette allocation. Par ailleurs, ce texte rappelle, dans ses motifs, l'importance, pour l'allocataire, de voir son autonomie assurée. Le groupe Union Centriste, au nom duquel je m'exprime cet après-midi, demeure pleinement attentif et sensible Il me vient en mémoire cette belle conclusion formulée par Sylvain Tesson dans une oeuvre récompensée en 2011 par un prix dont le nom résonne si particulièrement dans ces murs- je veux bien évidemment parler du prix Médicis Essai L'autonomie pratique et matérielle ne semble pas une conquête moins noble que l'autonomie spirituelle et intellectuelle. » Ainsi, comme l'ont précisé très justement ses auteurs, cette proposition de loi tend à améliorer la situation matérielle et morale de tout allocataire vivant en couple.

Les conséquences en termes d'unions sont avérées. C'est pourquoi l'article 1du texte vise à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans le versement de l'AAH quand celle-ci est versée en complément des autres ressources du bénéficiaire. 2 le prolonge en visant, cette fois, le plafonnement de l'aide financière. La baisse du coefficient de prise en compte des revenus du conjoint, à 1,8 au 1 janvier 2020, empêchera les allocataires vivant en couple de bénéficier pleinement de l'augmentation à 900 euros. ce tour de passe-passe comptable est choquant et critiquable. Cependant, il convient de préciser que d'autres minima sociaux, en lien ou non avec le handicap, prennent en compte les ressources du foyer. C'est notamment le cas du revenu de solidarité active. D'autres prennent même en considération le montant du patrimoine, par le biais des relevés de compte, comme l'aide personnalisée au logement. Par conséquent, si la question de la refonte se pose pour l'allocation aux adultes handicapés, elle demeure également légitime pour l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le revenu de solidarité outre-mer, l'allocation veuvage et tant d'autres encore. encore. Christophe Sirugue, dans un rapport remis au Gouvernement le 18 avril 2016, nous invite d'ailleurs à « clarifier l'architecture des minima sociaux » pour « renforcer son acceptabilité et fonder le consentement de tous à l'effort de solidarité Plus récemment, les rapports remis par Christine Cloarec-Le Nabour et Julien Damon, puis par Claire Pitollat et Mathieu Klein corroborent les besoins de rationalisation et de simplification des minima sociaux.

du problème. Il serait préférable d'envisager une réforme d'ensemble, plus complète, sur les différentes allocations. Nous nous devons d'impulser une politique qui s'inscrirait dans ce sens. C'est l'essence même des travaux de la Haute Assemblée.

Celui-ci est appelé à évoluer. Par corrélation, le budget finançant ces mesures le sera inéluctablement. Comme l'indique la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, dans une publication rendue publique le 15 octobre dernier, le nombre de bénéficiaires de l'allocation aux a doublé depuis 1990, pour atteindre 1,13 million de personnes à la fin de l'année 2017. Le contexte démographique et économique explique en partie cette considérable évolution. À cet égard, la présentation du mécanisme de financement soumis à notre approbation ne semble pas suffisamment convaincante. C'est pourquoi, même si nous soutenons l'esprit général du texte, nous appelons de nos voeux une réforme globale des minima sociaux, qui ne devra pas oublier la spécificité des personnes handicapées et qui pourrait réviser le mode de calcul de l'AAH. La solidarité devra être coordonnée avec les prestations de compensation.

Selon la proposition de loi de nos collègues du groupe CRCE, le titulaire de cette allocation doit pouvoir conserver ce revenu sans que soient prises en compte les ressources du conjoint ou de la famille. Il s'agit donc de désindexer cette aide sociale de l'État de la situation maritale de la personne handicapée. qui ouvre droit actuellement au versement mensuel d'une somme de 819 euros, fonctionne en intégrant les revenus du conjoint. Elle relève donc non pas d'une logique d'indemnisation, mais d'une logique de solidarité. Elle a été créée en 1975 par le gouvernement de Jacques Chirac.

n'est plus versée lorsque le conjoint perçoit plus de 2 200 euros. Le plancher de 1 126 euros, qui déclenche la dégressivité de l'AAH, et le plafond

Il est normal, dans le cadre de la solidarité, qu'il soit tenu compte des revenus du couple, tout en faisant évoluer le plancher et le plafond. Et pourquoi

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, il nous faut nous prononcer aujourd'hui sur une proposition de loi de notre collègue Laurence Cohen, qui vise à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés, aide financière accordée aux personnes atteintes d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ou compris entre 50 % et 79 % en cas de restriction durable d'accès à l'emploi ne pouvant être compensée par un aménagement de poste.

Pour mes collègues auteurs de la proposition de loi, la prise en compte des ressources du conjoint serait contraire au principe même de l'allocation, qui est de garantir l'autonomie du bénéficiaire. Elle instaurerait une relation de dépendance financière de l'allocataire à l'égard de son partenaire. Or, en réalité, l'AAH est destinée à compléter les autres ressources de la personne en situation de handicap et se cumule à d'autres aides qui sont, elles, individuelles, notamment le complément de ressources, ouvert pour chacun des membres du couple, la majoration pour la vie autonome, la pension d'invalidité et, éventuellement, le RSA. il convient de préciser que l'AAH est une prestation en espèces, et non en nature : elle vise à combler une perte de revenus. Or toute attribution de revenus en espèces, surtout dans le cadre des politiques de solidarité, est réalisée sur la base du foyer. L'AAH est donc un complément bien distinct de la PCH, laquelle est destinée à répondre, par une prestation en nature, aux dépenses liées à l'autonomie et aux besoins nés des difficultés de la vie quotidienne. Nous avons la chance d'avoir, en France, un système de solidarité comme il en existe rarement dans le monde, protégeant les plus vulnérables par l'effort national. Il faut en avoir conscience. Nous pouvons, animés de cet esprit, continuer de le parfaire. Il serait plus pertinent, à mon sens, de se pencher sur la PCH pour redéfinir ses périmètres et son montant, afin de l'adapter au mieux à notre société en mutation.

je considère que c'est la PCH qu'il serait logique et utile d'augmenter. De plus, la volonté de nier la situation familiale du bénéficiaire pour individualiser l'allocation, l'arracher à la dépendance financière de sa famille ou de son partenaire participe de cette vision individualiste de l'homme et de la société

par la loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement a prévu que les règles de prise en compte des revenus d'un couple percevant l'AAH seront rapprochées de celles qui sont appliquées aux autres bénéficiaires des minima sociaux, lesquelles sont bien moins avantageuses. Il s'agit là d'une manipulation purement technocratique. Par un savant calcul et par un jeu de balances, le plafond de ressources restera le même. L'augmentation de l'AAH n'aura donc strictement aucun impact sur les allocataires vivant en couple, ainsi que le rapport budgétaire de l'année dernière Quelle est donc cette mesure qui donne d'une main pour reprendre de l'autre ? Quelle est donc cette mesure qui permettra au Gouvernement de se vanter d'avoir augmenté une allocation alors que, en réalité, rien ne change pour une bonne partie des personnes concernées ? Quel est donc ce gouvernement qui utilise le handicap pour construire de fausses mesures non pas en faveur des bénéficiaires de cette allocation, mais dans son intérêt propre, en pensant sans aucun doute à son image ? cela ne s'arrête pas là : le Gouvernement a annoncé son souhait de supprimer le complément de ressources de 179 euros dont bénéficient les personnes handicapées à 80 % qui n'ont pas pu travailler depuis un an, à savoir les plus démunis.

a pour vocation de garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées ne disposant d'aucun revenu ou ayant de faibles revenus. Cette allocation est subsidiaire est subsidiaire : avant d'en demander le bénéfice, la personne handicapée doit faire prioritairement valoir ses droits, soit à l'invalidité, dans le cas de la pension d'invalidité, soit aux avantages vieillesse ce n'est que si les droits à l'assurance vieillesse ou à l'invalidité perçue par le demandeur se révèlent inférieurs au montant de l'AAH qu'elle pourra en bénéficier. Elle est différentielle : son montant s'ajuste aux autres revenus perçus par l'allocataire après divers abattements. Elle est familiarisée : elle tient compte de la composition du foyer de l'allocataire.

Doit-elle être considérée comme une aide individualisée ? C'est ce que suggère la proposition de loi du groupe CRCE, qui vise à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH,

Cette logique de solidarité nationale ou familiale s'articule aussi avec une logique de compensation, sans considération de ressources ou de foyer, et qui indemnise le préjudice subi par la personne handicapée. L'indemnisation est assurée par la prestation de compensation du handicap, la PCH, versée par les conseils départementaux, un dispositif situé hors du champ de la Pourrait ainsi se poser la question de savoir si l'AAH, qui fait partie des minima sociaux, devrait devenir une prestation compensatoire. Venons-en aux chiffres. Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le montant de l'AAH est passé de 810 euros à 819 euros au 1 avril 2018.

avec toutefois un coefficient de 1,9 pour l'AAH, contre 1,5 pour le RSA en 2018, et 1,8 en 2019. En d'autres termes, le montant de l'allocation a augmenté, mais le taux de cumul a diminué.

parcellaire et quelque peu réductrice, même si l'intention est évidemment louable. Reste à poursuivre le chantier engagé sur la question plus générale des minima sociaux et la réflexion sur la reconnaissance de la spécificité de l'AAH telle que voulue, par exemple, par l'Association des paralysés de France. Reste Reste au-delà à mettre en oeuvre une véritable réflexion sur la place des personnes handicapées, en particulier les personnes handicapées vieillissantes, sans doute les plus démunies ; selon moi, elles devraient bénéficier de structures d'accueil spécifiques. Reste enfin, dans le cadre de la refonte des minima sociaux autour peut-être du revenu universel d'activité, à réfléchir à la notion de minima sociaux différenciés en fonction de critères objectifs selon l'âge, les territoires, le statut des bénéficiaires.

notre groupe a fait le choix de déposer au Sénat la proposition de loi qui a été portée à l'Assemblée nationale par notre amie et collègue députée Marie-George Buffet, du groupe Gauche démocrate et républicaine. le texte a été cosigné par des députés issus de groupes politiques extrêmement divers, allant des Républicains à la France insoumise, en passant par l'UDI, le Modem et les socialistes ; il a même été signé par des députés du groupe La République En Marche.

Alors qu'il y avait à l'évidence un large rassemblement sur le sujet, nous avons été surpris et déçus par le vote négatif de la commission des affaires sociales du Sénat sur notre proposition de loi, dont l'auteur est mon amie Laurence Cohen. Cohen. Nous avons bien entendu les arguments de la majorité sénatoriale, qui reproche notamment le coût de la mesure et préférerait une refonte complète de l'ensemble des dispositifs existants, au lieu de se limiter, comme nous le proposons, à la suppression de la prise en compte des revenus des conjoints dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Mes chers collègues, oui, notre proposition de loi a un coût ! Oui, une réforme globale des aides sociales pour lutter contre le non-recours est indispensable Mais notre objectif est avant tout d'envoyer un signe positif aux personnes en situation de handicap, qui, malheureusement, se sentent trop souvent rejetées et regardées comme des citoyens de seconde zone Il faut remettre de l'humain au coeur des décisions politiques et en finir avec le sentiment de mépris que subissent les personnes en situation de handicap, auxquelles on a promis l'égalité en 2005. Nous devons faire un geste pour leur rendre la dignité qui leur est due. Le Président de la République a effectivement dit que le handicap était une priorité de son quinquennat. Mais, au-delà des paroles, il faut passer aux actes. Après l'annonce de la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés à 900 euros à grand renfort de communication par le Gouvernement, les personnes handicapées- faut-il le rappeler ? -ont subi depuis un an une série de reculs suppression du complément de ressources au 1 janvier 2019, soit 179 euros en moins chaque mois pour les futurs allocataires ; baisse de l'obligation de 100 % à 20 % de logements neufs accessibles dans la loi ÉLAN suppression de la prise en charge des sorties thérapeutiques pour les personnes rejoignant leur famille le week-end. À ces mesures spécifiques aux personnes en situation de handicap, il faut encore ajouter la baisse des APL, la hausse de la CSG, la désindexation des pensions de retraite, qui concernent tous les Français.

La Haute Assemblée doit envoyer un signe positif en supprimant l'injustice qui consiste à prendre en compte dans un couple les revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. C'est une question de respect de la dignité des personnes que d'accorder cette allocation à l'ensemble des hommes et des femmes qui ont un taux d'incapacité supérieur à 80 %. si le conjoint a des revenus supérieurs à 1 126 euros, le montant de l'AAH devient dégressif. Si les revenus sont supérieurs à 2 200 euros par mois, l'AAH n'est plus versée aux allocataires.

Hémiplégique gauche depuis dix ans, elle n'a le droit ni à la pension d'invalidité ni à l'allocation aux adultes handicapés, car son mari a des revenus supérieurs aux critères, ce qui la met dans une situation de dépendance vis-à-vis de lui. Publié par l'Association des paralysés de France, le témoignage de Marie vient rappeler que des personnes handicapées se retrouvent privées d'aides et donc dépendantes financièrement de leur conjoint à l'âge de soixante soixante ans. Le cas de Marie n'est pas un cas isolé, et vous le savez : nous avons tous autour de nous des personnes handicapées qui ne peuvent compter que sur l'aide des familles pour payer leur loyer, leurs frais de santé ou leurs courses, car la solidarité nationale est défaillante. Sans la solidarité familiale, les individus seraient dans l'incapacité de faire face aux démarches du quotidien. Madame la secrétaire d'État, l'État doit prendre ses responsabilités et s'engager en faveur des personnes handicapées pour garantir des conditions de vie dignes. Mes chers collègues,

les associations, les fédérations d'associations et d'employeurs, y compris le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Il est à craindre que les mesures de revalorisation, promesse de campagne du Président du Président de la République, ne se heurtent à des réalités budgétaires non anticipées. Les rapporteurs spéciaux ont en effet souligné que l'AAH n'était pas un minimum social comme les autres. Si ce débat concerne

de mai dernier, j'attirais l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'indispensable modification des règles de calcul pour l'attribution de l'AAH, qui pénalisent les personnes en situation de handicap vivant en couple dès lors que les revenus du conjoint dépassent 1 126 euros mensuels et qui conduisent à la suppression de l'AAH dès que les revenus du conjoint atteignent 2 252 euros mensuels. La réponse apportée était loin de me satisfaire, puisqu'il était indiqué qu'à l'occasion de la revalorisation exceptionnelle de l'AAH à 860 euros le 1 novembre 2018 le coefficient multiplicateur passerait à 190 %, puis à 180 % le 1 novembre 2019 lors de la seconde hausse à 900 euros. En clair, la baisse du coefficient multiplicateur compense la hausse du plafond pour une personne seule, l'objectif étant de rapprocher les règles entre minima sociaux. Cela renforce ni plus ni moins la dépendance financière dans laquelle sont maintenues les personnes en situation de handicap à l'égard de leur conjoint, ce qui est inacceptable et honteux ! Ainsi, 250 000 allocataires en couple ne vont pas bénéficier du gain de 90 euros qu'a fait miroiter le candidat Macron, ce qui permettra au Gouvernement d'économiser en moyenne 450 millions d'euros par an, soit 80 % du coût de l'augmentation de l'AAH, estimée à 550 millions d'euros en année pleine. De même, pouvez-vous nous indiquer, madame la secrétaire d'État, le devenir du complément de ressources dont bénéficient 65 000 personnes environ, soit 6 % des allocataires ? S'il devait disparaître au profit de la majoration pour la vie autonome, ce qui reviendrait à conserver le complément le moins avantageux, ce serait un coup de massue supplémentaire pour les allocataires lourdement handicapés, qui perdraient une partie de la hausse promise par le candidat Macron ! Pour toutes ces raisons, de loi est vitale pour nos concitoyens atteints d'un handicap, auxquels nous nous devons d'apporter des gages de sécurité financière au nom de la justice sociale. La parole

ne soutiennent pas une telle initiative. D'ailleurs, on les sent relativement embarrassés. Quand on discute sur le fond, ils trouvent assez juste que le principe de dignité et d'autonomie des personnes soit affirmé

que chaque personne apporte quelque chose. L'autonomie des personnes handicapées est une question majeure pour notre projet de société. Et l'effort financier demandé est dérisoire au regard de bien d'autres cadeaux fiscaux beaucoup moins utiles

du seul fait de la suppression d'un plafond doublé. Je vous le rappelle, quel que soit le plafond de ressources, le montant individuel de l'AAH ne peut pas dépasser le plafond individuel, même lorsque le bénéficiaire est en couple.

structuré, de l'aveu même du Gouvernement, autour de l'ambition « d'accélérer la baisse du déficit public et des prélèvements obligatoires »- et de porter, au nom de cet objectif, un nouveau coup à notre modèle social

C'est avec la dette publique que nous avons reconstruit nos routes et nos ports, développé notre réseau autoroutier, nos aéroports internationaux ! C'est avec la dette publique que, devant la pénurie de logements, nous avons créé notre patrimoine locatif social, réponse pertinente au mal-logement C'est avec la dette publique que nous avons réalisé, en même temps que se généralisait la sécurité sociale, l'équipement du pays en hôpitaux de haut niveau, qui participent encore de nos atouts C'est avec la dette publique que nous avons pu mettre à l'étude la fusée Ariane, avant d'en faire l'un des meilleurs lanceurs de satellites de la planète ! C'est avec la dette publique que nous avons lancé les études qui ont conduit à la conception du TGV dit, chaque fois que le besoin s'en est fait sentir, chaque fois que l'attractivité et les conditions de développement de notre pays l'ont exigé, nous avons su utiliser l'outil de la dette publique pour créer les conditions d'une avancée supplémentaire pour notre pays, pour son économie, pour sa société

C'est avec la dette publique que les collectivités territoriales prennent aujourd'hui en compte les équilibres écologiques, protègent les zones naturelles sensibles, développent les transports publics. Mais, comme vous le savez, mes chers collègues, c'est aussi avec la dette publique que nous avons, dans le passé, payé la lourde facture des aventures militaires coloniales C'est avec la dette publique que nous avons payé et que nous payons encore le prix des restructurations économiques, des plans de licenciement, des réductions d'impôt sans pertinence, des allégements de cotisations sociales riches d'effets pervers, des déficits publics consentis au nom de la compétitivité.

les taux d'intérêt se sont réduits, et noterons, pour notre part, que l'inflation semble bien avoir consommé une part essentielle de ce qui a été regagné sur ce que j'appelle, quant à moi, le « loyer de l'argent ». Toujours est-il que, dette publique ou dette privée, il semble bien que nous ayons hérité de la nécessité de les souscrire,

un État, s'endetter auprès des marchés financiers -insistons sur ce point, car c'est à eux que vont les 43 milliards d'euros d'intérêts inscrits au budget de l'État -parce qu'il a renoncé à des recettes fiscales essentielles

il y avait une dette publique, ne serait-ce que parce qu'il est toujours bienvenu de proposer un produit d'épargne sécurisé au grand public ; le marché boursier était alors largement dominé par les échanges de titres obligataires.

Prenons l'exemple du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, l'une des mesures phares du quinquennat Hollande, que l'on s'apprête aujourd'hui à transformer en allégement pérenne de cotisations sociales, ce qui ne me semble guère pertinent.

Mais comment ne pas souligner que, pour éponger la facture, on a aussi relevé les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui a porté atteinte au pouvoir d'achat des ménages, ainsi qu'à la capacité d'autofinancement des collectivités locales des collectivités locales ? Celles-ci n'ont-elles pas payé, au fil des ans, le prix du CICE la remise en cause du montant de leurs dotations, et singulièrement de la dotation globale de fonctionnement ? La question est posée.

Mais ce qui fait le plus mal, mes chers collègues, ce sont les 55 milliards d'euros de dotation globale de fonctionnement perdus en cumulé depuis 2012.

Le rapport du comité de suivi est plus prudent : « Le comité maintient les conclusions avancées dans les précédents rapports et retient un effet net qui serait proche de 100 000 emplois créés ou sauvegardés et qui se serait matérialisé sur 2014 et 2015 dans les entreprises les plus exposées au CICE. Le comité tient pour robustes les résultats des équipes qui concluent à un effet positif du CICE sur les salaires moyens et la masse salariale. Toutefois, aucun effet du CICE sur les salaires au niveau individuel n'est identifié à proximité du seuil de 2,5 SMIC, sur les salaires d'embauche comme sur les augmentations salariales des employés permanents. « Le comité constate que l'existence d'un effet significatif du CICE sur l'investissement demeure difficile à établir sur la période 2013-2015. » Nous avons là la démonstration systémique des effets que peut produire un vecteur essentiel de dette publique. Cet exemple est probant, puisqu'il y va de l'abandon d'une recette fiscale de plus de 80 milliards d'euros au titre de l'impôt sur les sociétés et d'un peu plus de 4 milliards d'euros au titre de l'impôt sur le revenu.

Revenons d'ailleurs sur le cas des ménages : pourquoi leur taux d'endettement connaît-il ces derniers temps une hausse relative, alors que tel n'est pas le cas dans la zone euro en général ? La hausse de la production de prêts immobiliers, liée à la détente des taux d'intérêt, explique sans doute en partie le phénomène, sans parler des modalités fortement incitatives d'achat de véhicules, avec la pratique du crédit par loyer mensuel. l'endettement signifie aussi, dans ce contexte, insuffisance de revenu et d'épargne. On ne doit, en l'espèce, jamais oublier que ce sont les segments divers de l'endettement privé qui ont mené, ces dernières décennies, les économies occidentales à la crise financière,

assorti d'une période de récession source de chômage et de déficits publics ; explosion de la dette publique, dans le second cas, avec une nouvelle récession dont nous ne sommes toujours pas rétablis. Nous ouvrons aujourd'hui le débat pour que chacun puisse donner son avis,

soit une dette réelle dépassant les 6 000 milliards d'euros ! Ces engagements hors bilan sont un véritable fourre-tout, dans lequel les gouvernements successifs ont entassé les sommes qu'ils anticipaient devoir payer un jour, sans réellement s'en soucier.

Depuis trop longtemps, la réduction de la dette est une chimère dans notre pays. En effet, nombreux sont les gouvernements ayant juré, la main sur le coeur, de s'attaquer à la diminution de la dette. Mais aucun ne s'y est effectivement attaché. Très rares sont les résultats, mais abondants sont les rendez-vous manqués, les excuses démagogiques et les lâchetés. C'est cette lâcheté qui coûtera cher aux générations futures. Certains pensent que l'État ne se gère pas comme une entreprise ; tel n'est pas mon cas. Qu'ils sachent que l'histoire montre qu'une dette est une dette, et que les cigales finissent toujours par passer à la caisse. J'ai bien sûr conscience qu'il y a une bonne et une mauvaise dette. La bonne dette, c'est celle qui soutient l'investissement, l'innovation, et qui est à l'origine de la richesse de demain. juste ! La mauvaise dette, c'est celle qui sert à financer le fonctionnement d'un État trop lourd et trop peu efficace. Or, aujourd'hui, c'est encore largement la mauvaise dette qui domine en France, et qui ne recule jamais tout à fait.

Sans grande réforme de l'action publique, nous n'aurons que des budgets au fil de l'eau nous éloignant de l'efficience et nous plongeant chaque fois plus profondément dans une insouciance trompeuse. J'ai ainsi le regret de constater, monsieur le secrétaire d'État, que nous sommes encore bien loin d'un État moderne, c'est-à-dire d'un État modeste

soit presque autant que le budget de l'éducation nationale. Vous conviendrez que cela ne correspond pas tout à fait à ce que l'on pourrait appeler un « investissement d'avenir » ! Cet argent va aux marchés financiers que mes collègues de gauche adorent

d'ailleurs de relever ses taux après l'été 2019, ce qui aura pour conséquence de fragiliser la situation des pays de la zone euro particulièrement endettés.

vu ! Monsieur le secrétaire d'État, eu égard à ces éléments, quelle sera la facture de votre héritage pour les générations futures ? Il y a quelques mois, vous vouliez changer le monde politique : commencez par changer les politiques budgétaires ! Si vous voulez vraiment une France en marche, faites que l'État ne marche plus sur la dette

On parle souvent du fardeau qu'elle représente pour les générations futures : c'est une réalité, mais je m'inquiète également du déclassement économique dont elle menace la France. Tous nos voisins européens ont entrepris un désendettement vigoureux, notamment l'Allemagne. Le différentiel d'endettement avec ce pays atteindra bientôt 39 points de PIB : cette situation est inédite dans l'histoire récente. Comment espérer peser politiquement en Europe sans être exemplaire ? Comment espérer entraîner nos partenaires en demeurant « l'homme malade de l'Europe » ? Le désendettement de notre pays est une priorité politique. Le une priorité pour préserver notre souveraineté. Quand la dette atteint 100 % du PIB, une remontée des taux d'intérêt représente un danger de premier ordre pour le budget de l'État. Le service de la dette est déjà le deuxième poste de dépenses de l'État ; il pèse soit cinq fois plus lourd que le budget de la justice. Cette situation inadmissible pourrait vite devenir insoutenable dans un contexte de hausse des taux : selon l'Agence France Trésor, une remontée de 200 points de base des taux d'intérêt ferait presque doubler la charge de la dette. En l'absence d'une politique de consolidation budgétaire, la hausse de la charge de la dette pourrait ainsi atteindre des proportions incontrôlables. Cet enjeu conditionne donc la viabilité de nos finances publiques. deuxième urgence est celle de l'instabilité financière : je veux parler des risques que fait peser sur notre économie la dette privée. La dette des entreprises et des ménages atteignait 130 % du PIB en 2017. En 2007, juste avant le début de la crise financière internationale, elle était encore légèrement en dessous de 100 % du PIB. N'oublions pas que la crise financière de 2008 est une crise de la dette privée avant d'être une crise de la dette publique Certes, nous avons renforcé la régulation prudentielle aux niveaux national et européen depuis 2008. Mais les politiques monétaires accommodantes, la hausse des prix de l'immobilier et le retour de la croissance font peser des risques sur cet endettement. Je déplore que plusieurs voix, aux États-Unis et en Europe, appellent à une moindre régulation financière, au démantèlement des institutions et des normes que nous avons mises en place. Il faut, au contraire, continuer à s'engager pour une finance plus saine, plus responsable et mieux encadrée. Cet engagement n'a de sens qu'au niveau européen : nous appelons à l'achèvement de l'union bancaire et de l'union des marchés de capitaux, qui permettra de maîtriser l'endettement et de prévenir les crises. Enfin, la dernière urgence, fortement liée aux deux autres, est celle de la volonté politique. Nous devons rompre avec un État dopé à la dépense publique : il y va de la préservation de notre souveraineté nationale et de notre mode de vie. Je crois profondément que cette question sera le juge de paix du quinquennat d'Emmanuel Macron. force est de constater que nous n'y arrivons pas. Nous multiplions les revues de dépenses, les comités, les rapports, mais la dépense publique ne baisse pas, ou si peu. La logique budgétaire n'a pas basculé d'une logique de moyens vers une logique de résultats. Le nombre de fonctionnaires diminue trop lentement pour que les objectifs fixés par le Président de la République puissent être atteints. Bref, les conditions ne sont pas réunies pour une diminution ambitieuse de la dépense publique qui permette un désendettement rapide. Je souhaiterais terminer, monsieur le secrétaire d'État, en vous réitérant le soutien du groupe Les Indépendants à votre entreprise de diminution de la dépense publique. Il s'agit d'une question d'intérêt national qui appelle une union sacrée. C'est la responsabilité de notre génération de lever cette hypothèque qui pèse sur l'avenir du pays et sur celui de nos enfants.

La dette publique n'est pas, contrairement à ce que peuvent peut-être penser nos collègues du groupe CRCE, dictée par les marchés ou la technocratie de Bruxelles pour faire accepter des sacrifices au peuple. Elle est le résultat de l'inconséquence budgétaire des gouvernements qui se qui se sont succédé depuis la fin des années soixante-dix. Faire fi de la dette va à l'encontre du bon sens populaire. C'est la cigale de la fable de La Fontaine qui, n'ayant cessé de dépenser sans compter, se trouva fort dépourvue quand la crise fut venue Chaque Français comprend bien que l'on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on gagne, sauf à emprunter pour investir. Or la part des dépenses d'investissement dans les dépenses publiques n'est aujourd'hui que de 6 %, ce qui signifie que la dette française ne crée pas de valeur, ou très peu. La France dépense 280 milliards d'euros de plus que l'Allemagne et est depuis 2016 la championne d'Europe de la dépense publique Ce niveau de dépense publique nous rend dépendants de notre niveau de recettes. Sans hausse de la fiscalité ou retour de la croissance, il n'est pas possible de diminuer notre déficit public et notre dette. Or nous n'avons plus de marges de manoeuvre sur les recettes, la France étant également championne d'Europe des prélèvements obligatoires, sans pour autant que son niveau de recettes couvre son niveau de dépenses.

la préoccupation du groupe CRCE. Notre collègue Éric Bocquet a mis en évidence l'importance du phénomène dans ses différents rapports. Un dernier scandale est venu illustrer l'ampleur de la fraude les États européens auraient été floués à hauteur de 55 milliards d'euros par an pendant quinze ans, la France de 3 milliards d'euros chaque année. Mais la lutte contre la fraude fiscale ne suffit pas.

si l'on tient compte de l'intégration de la dette de SNCF Réseau dans les comptes publics. Ce manque d'efforts n'est pas nouveau : soit les gouvernements ont laissé filer les déficits, soit ils ont subi des crises qui ont accéléré l'endettement.

Malgré des taux d'intérêt extrêmement bas actuellement, la charge de la dette représente le deuxième budget de l'État après celui de l'enseignement scolaire, avec plus de 41 milliards d'euros en 2018, soit plus du double du budget alloué à la sécurité

la Banque de France s'inquiète de l'endettement des entreprises, qui ne cesse d'augmenter : en mars 2018, cette dette représentait près de 73 % du PIB, contre 60 % en moyenne dans la De la même façon, la dynamique de l'endettement des ménages, notamment celle des crédits immobiliers, est forte. Pour le Haut Conseil de stabilité financière, son niveau justifie une « vigilance renforcée ». En cette période où les risques de crise systémique n'ont pas disparu, rappelons-nous que la crise des avait ruiné nombre d'Américains, les poussant à vendre leur maison. Car, à la différence de la dette publique, la dette privée sert à financer des biens. En cas de crise, l'emprunteur privé n'a d'autre solution que de les liquider. L'excès de crédit à la consommation aux États-Unis, la bulle immobilière en Suède et au Canada, la bulle des crédits aux économies émergentes et la situation actuelle en Italie sont autant de risques économiques potentiels. Il convient donc d'agir à tous les niveaux pour réduire l'endettement privé et public, avant qu'une nouvelle crise d'ampleur ne survienne et ne crée une spirale négative qui pourrait être mortifère. Ayons donc le courage, au regard de ces vérités, de réduire la dette, publique et privée, que supportent les Français et qui bride nos capacités d'investissement. Il y a urgence

du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics. J'y vois une structuration intelligente pour transformer durablement l'administration, qui vient prolonger la création d'un fonds de transformation de l'action publique. À la demande du groupe CRCE, le Sénat est invité à s'exprimer sur la dette publique et la dette privée. En 2017, la dette des administrations publiques a représenté 98,5 % du PIB en 2018, elle devrait atteindre 98,7 % du PIB. Cette dette publique correspond au montant que les Français souhaitent dépenser pour bénéficier d'un certain niveau de service public. Dit autrement, en l'absence de transferts internationaux, les dépenses publiques sont financées par l'impôt, c'est-à-dire les contribuables d'aujourd'hui, ou par l'emprunt public, c'est-à-dire les contribuables de demain. L'emprunt consiste en des titres de créance vendus par l'État à des investisseurs, donnant droit à des versements en capital et en intérêts. Aujourd'hui, la charge des intérêts de la dette de l'État, inscrite au programme 117

Un niveau élevé de dette publique n'est pas propre à la France. Dans les pays développés, l'encours de la dette publique a quasiment doublé entre 2007 et 2017, passant de 71 % à 105 % du PIB. Cette forte évolution consécutive à la crise de 2007 a joué le rôle de stabilisateur macroéconomique, la relance budgétaire ayant été concertée entre les pays du G20 et efficace. Cela doit nous rappeler une évidence en matière de politique économique

Autrement dit, la France a les mains liées pour faire face au choc qui arrive. Les risques liés à un niveau de dette publique élevé sont bien définis par les néoclassiques. Une étude récente du CEPR, le Centre for Economic Policy Research, basé à Londres, met en évidence une corrélation négative entre la dette publique et l'investissement des entreprises un niveau élevé de dette publique est associé à un plus faible investissement privé. Depuis la crise, le montant de la dette mondiale, publique et privée, a progressé, sous l'effet de la contraction de l'activité et de pressions déflationnistes.

La question du niveau d'endettement ne doit être posée qu'au regard des dépenses financées ; les entreprises et les ménages ont pu profiter des taux extrêmement bas pour financer des investissements. Pour autant, des motifs d'inquiétude existent. Ainsi, dans son bulletin trimestriel de septembre dernier, la Banque des règlements internationaux met en lumière les risques liés à des conditions faibles et à des bilans de banques anormalement élevés. La situation financière doit retenir notre attention.

nécessité de diminuer l'endettement public et celle de mettre en place une surveillance accrue au niveau européen. Sur le premier point, le Gouvernement et la majorité présidentielle se sont engagés sur une trajectoire de réduction des dépenses publiques. Pour la première fois

Bien que cela paraisse difficile à croire, un tel effort est inédit. C'est la première fois que la dépense est sous 1 % trois fois de suite et c'est la plus grande baisse de la dépense publique depuis cinq quinquennats.

La crise espagnole était, quant à elle, financière et immobilière : la baisse des taux d'intérêt a favorisé des investissements non productifs et la formation d'une bulle immobilière. Face à cela, la conduite de la politique économique espagnole n'a pas été équilibrée. Certes, depuis la crise, la surveillance budgétaire en Europe a été renforcée, avec le six-pack, le two-pack et le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui encadre fortement les finances publiques des États membres. Mais les efforts de convergence des marchés européens doivent être accentués. Par ailleurs, pour mieux accompagner les chocs et les bas de cycle, une assurance fédérale pourrait être mise en place. Cela permettrait d'envoyer un signe fort aux populistes. Pensons par exemple à un système européen d'assurance chômage qui reposerait sur un préalable

En effet, depuis plusieurs décennies, la dette publique est devenue la clef de voûte des exercices budgétaires des différents gouvernements. Le discours répété à l'envi par des dirigeants successifs est le suivant : la France vit au-dessus de ses moyens, si nous ne faisons rien les marchés financiers vont nous punir en augmentant les taux d'intérêt, ce qui renchérira le coût de l'emprunt et accroîtra encore plus notre dette ; cette fuite en avant risque de nous mener tout droit vers la faillite et ce seront les générations futures qui devront rembourser nos excès. Tel est le discours officiel constamment répété par les gouvernements. ce discours mérite un examen un peu plus attentif. Est-il pertinent de comparer la dette d'un pays à celle d'un ménage, comme cela se fait couramment ? Un pays ne meurt pas et ne peut être saisi.

Lorsque l'on dit que la dette représente 100 % du PIB, on compare une dette, dont le remboursement s'échelonne sur plusieurs années, à une valeur annuelle, le PIB. Cela n'est jamais le cas pour un ménage. Si l'on applique le même mode de calcul à un couple gagnant 32 000 euros par an et ayant une dette de 200 000 euros liée à l'achat d'un appartement remboursable sur de ce ménage représente 625 % de ses revenus d'activité. On en conviendra, une telle situation est vécue par bon nombre de nos concitoyens. Pourquoi la Commission européenne, si prompte à inciter les pays à appliquer des mesures d'austérité, ne condamne-t-elle pas les paradis fiscaux en Europe, permet à plusieurs dizaines de milliards d'euros d'échapper au budget de la République ? Le budget de la France n'a plus été équilibré depuis 1973, soit quarante-quatre années de déficits cumulés. Le 3 janvier 1973, il fut décidé par les gouvernants de l'époque que l'État pourrait se financer auprès des marchés financiers et non plus auprès de la Banque de France. Puis vint le traité de Maastricht, en 1992. Aux termes de son article 104, « il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées " banques centrales nationales ", d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions

ceux qui gèrent l'épargne des retraités américains ou britanniques, ensuite les fonds mutuels ou sociétés d'investissement et, enfin, les compagnies d'assurances et les banques, y compris françaises.

Les économistes bien en cour, orthodoxes, nous expliquent régulièrement que la dette serait causée par une prétendue incurie et gabegie de l'État. Pourtant, quand on examine très précisément les chiffres, les dépenses publiques restent, en proportion, assez stables depuis de nombreuses années. C'est bien évidemment d'un déficit de recettes que nous pâtissons essentiellement. Pour notre part, nous pensons qu'il y aurait lieu de procéder à un audit sérieux et intégral de notre dette publique. En quarante ans, la France a déjà payé plus de 1 400 milliards d'euros d'intérêts à ses créanciers. Il faudrait bien sûr évaluer l'impact des multiples dégrèvements, abattements, exonérations et autres crédits d'impôt, qui se sont chiffrés en dizaines de milliards d'euros depuis une vingtaine d'années. Il y a aussi bien sûr l'enjeu de la lutte contre l'évasion fiscale. Nous posons la question : quelle est, dans le total, la part de dette légitime ? Si, au lieu de se financer depuis trente ans sur les marchés financiers, l'État avait contracté des emprunts directement auprès des ménages ou des banques, à des taux d'intérêt réels de 2 %, la dette publique serait aujourd'hui inférieure de vingt-neuf points de PIB, soit de 589 milliards d'euros, par rapport à son niveau actuel. Maurice Allais disait que « la création monétaire doit relever de l'État et de l'État seul ». La Banque centrale européenne ne devrait-elle pas jouer ce rôle économique essentiel, prêter aux États à taux faible plutôt que d'inonder les marchés financiers de liquidités énormes qui ne servent que très peu l'économie réelle ?

Vous le voyez, nous avons abordé dans ce débat les aspects financiers et budgétaires, bien sûr, mais aussi les questions de souveraineté, de démocratie et de liberté. Le philosophe Gilles Deleuze disait que « l'homme n'est plus l'homme enfermé mais l'homme endetté ». La parole

En effet, depuis plusieurs années, on entend dire que la dette publique serait l'une des causes, sinon la cause principale, de nos maux. Nous n'aurions plus les moyens d'assurer notre train de vie et il nous faudrait donc réaliser des économies au plus vite, nous vivrions au-dessus de nos moyens, ce qui freinerait les dynamiques économiques et ferait courir un risque aux générations futures, auxquelles nous léguerions comme héritage une dette lourde et injuste. Qu'en est-il exactement ?

il reste toutefois assez nettement inférieur à celui que l'on constate aux États-Unis- 149 % du PIB -, au Japon -147 % -ou au Royaume-Uni- 156 %.

-, comme l'un des critères privilégiés d'appréciation de la solvabilité des États. Néanmoins, certains analystes considèrent qu'il est discutable de comparer un stock, la dette, à un flux, le PIB, c'est-à-dire la richesse créée annuellement. Il paraît plus pertinent de mettre en regard la dette publique et le patrimoine public ; à cet égard, il faut noter une véritable lacune dans la connaissance des actifs de l'État.

Deuxièmement, la dette publique est sans cesse ramenée à une seule année de production annuelle, alors qu'il s'agit d'un engagement qui a vocation à être apuré sur plusieurs années. Enfin, l'approche patrimoniale des ménages ne peut être valablement appliquée à la gestion des comptes de l'État. La dette de l'État sert à financer ses interventions -infrastructures,

Il est important de considérer combien la dette est salutaire pour les classes moyennes et les plus pauvres, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une autre protection et d'autres services que ceux qui sont assurés par le service public. Grâce aux transferts sociaux, le taux d'enfants vivant dans une famille pauvre passe de 25 % à 8 %, le taux de pauvreté chez les retraités est en France l'un des plus faibles au monde, se trouvant réduit de quatre points par rapport à ce qu'il serait sans cette redistribution. Globalement, les transferts sociaux et fiscaux diminuent le taux de pauvreté monétaire de huit points. La France se situe ainsi parmi les pays où la redistribution sociale est le plus élevée. Ce n'est pas un problème, c'est clairement une solution. Enfin, à ceux qui véhiculent l'idée selon laquelle la dépense publique ne servirait qu'à financer le paiement des fonctionnaires improductifs, il faut répondre que, bien au contraire, les fonctionnaires contribuent au PIB : leur valeur ajoutée est estimée à 333 milliards d'euros, ce qui représente un tiers de celle des salariés des entreprises de droit privé. privé. La dette publique reflète précisément la place que l'État tient dans la société. Historiquement, la France est attachée à l'intervention de l'État dans les domaines régaliens, mais aussi dans les secteurs

C'est aussi cette histoire qui fait que la France figure aujourd'hui au sixième rang des puissances mondiales ; la place de l'intervention publique n'est un frein ni à sa compétitivité ni à son attractivité. Vous l'aurez compris, la dette publique engendre de la valeur ajoutée et de l'emploi. Elle permet de réaliser des infrastructures- routes, voies ferrées -et d'assurer des services- éducation, formation, santé -, autant de facteurs participant à la performance économique du pays. En témoigne notre attractivité, des dernières années, en matière d'investissements étrangers portant, notamment, sur des fonctions stratégiques telles que les centres de recherche et développement La dette publique permet de constituer le patrimoine de ceux qui n'ont pas, en mettant à disposition des infrastructures et des services assurant un traitement égalitaire en matière d'accès aux services publics,

augmenté, au cours des dernières années, leur dette publique, afin que le système ne s'effondre pas. Ils ont ainsi pu éviter que la grande récession ne se transforme en grande dépression.

la libéralisation financière, le libre-échange, l'austérité salariale et la contre-révolution fiscale, avec l'idée que les riches doivent payer moins d'impôts pour favoriser la création de richesse, laquelle doit, selon la théorie du ruissellement, profiter à tous. Ces dernières années l'ont montré, cela ne marche pas. Pis, la concentration de la richesse est de plus en plus grande, les disparités explosent et la pauvreté s'accroît. Le néolibéralisme a donc encouragé l'endettement privé, car, faute d'augmentations de salaire, les ménages ont dû emprunter

en Europe. Cette contre-offensive a été particulièrement forte ; il en est résulté l'impasse complète que nous subissons aujourd'hui : la baisse des dépenses publiques provoque la stagnation du chômage et de la croissance, et donc réduit les recettes fiscales. De ce fait, le déficit public ne se réduit pas, ou Les grandes institutions financières, FMI en tête, qui ont imposé cette austérité brutale en Europe et ailleurs reconnaissent désormais les effets négatifs d'une trop forte réduction de la dépense publique.

du pays. Nous devons impérativement faire porter nos efforts sur la dette privée, car, en vue de sortir de la crise financière, il convient désormais de s'interroger sur la libéralisation financière, le libre-échange, l'austérité salariale et la contre-révolution fiscale. il nous faut recréer au plus vite les conditions d'un véritable revirement des politiques à l'échelle européenne, en mettant au premier plan non plus l'austérité et la flexibilité, mais la relance sociale et les transitions économiques et écologiques. Il y a urgence ! La parole

par l'INSEE. En 2019, comme en 2018, l'État empruntera le montant record de 195 milliards d'euros sur les marchés.

Une fenêtre d'opportunité se présentait pour engager des réformes structurelles. Quelle est, à l'aune de telles considérations, la tendance actuelle ? La Banque postale prévoit une remontée du taux des obligations

conduirait à aggraver la charge de la dette de 2,1 milliards d'euros en un an, de 4,8 milliards d'euros en deux ans et de plus de 19 milliards d'euros en dix ans. Certes, nous pouvons toujours trouver un motif d'apaisement, ne serait-ce que temporaire, dans le fait que le taux de l'OAT à dix ans s'établit aujourd'hui autour de 0,80 %.

des non-résidents a fortement crû, passant de 28 % à la fin de 1999 à 67 % en 2010, avant de diminuer de façon marquée depuis la fin des années 2000.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, si la dette publique et la dette privée, des ménages et des entreprises, sont des sujets de grande préoccupation pour le Sénat, nos concitoyens eux-mêmes s'interrogent et s'inquiètent en constatant la dégradation continue des prévisions de déficit public pour les années à venir et leurs conséquences sur leur pouvoir d'achat et sur l'emploi. L'absence, dans les projets du Gouvernement, de véritables mesures structurelles permettant de réduire réellement la dépense publique renforce cette inquiétude. La dépense va encore alimenter la dette publique et réduire, une fois de plus, nos marges de manoeuvre. Le service de la dette, qui avoisine 50 milliards d'euros, est l'un des premiers postes du budget de l'État. D'aucuns prétendent que l'endettement de la France n'est finalement pas aussi grave au regard des actifs que l'on peut mettre en face, et, dans cette perspective, ils ratissent très large, mélangeant allègrement actifs publics et actifs privés, en oubliant que l'État est au service des citoyens, et non l'inverse. Envisager la dette comme une nécessité est une erreur profonde ! Il s'agit, au contraire, d'un dangereux héritage qui pèse sur l'ensemble des Français. Le déficit public s'élèvera à 2,6 % du PIB en 2018

Par ailleurs, le changement de politique de la Banque centrale européenne et l'arrêt de son programme d'achat d'actifs, qui a une incidence bénéfique sur les taux d'intérêt, peuvent avoir des conséquences négatives sur la notation de la France et la qualité de sa signature, surtout lorsque l'on sait, ou plutôt lorsque l'on ne sait pas,

La dette des ménages s'élève à 1 163 milliards d'euros, celle des entreprises non financières à 2 187 milliards d'euros. C'est un volume colossal, dont l'expansion a été favorisée par des taux d'intérêt artificiellement bas.

Pour désagréable que cela soit, il faut être réaliste ; les chiffres sont têtus ! Notre économie est financièrement fragile, et nos faiblesses en termes de compétitivité se traduisent dans le déficit de notre commerce extérieur. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie par avance des réponses que vous pourrez apporter à nos interrogations, qui sont également celles de nos concitoyens.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le thème abordé mériterait au minimum un rapport d'information, voire une thèse universitaire,

Pour l'héritage, on n'a pas le choix, sauf à envisager, comme certains ont pu le faire, de refuser de rembourser nos dettes au système bancaire, dont la légitimité serait contestée.

elle doit être assortie de considérations sur l'utilisation, le niveau, la gestion et les limites de la dette. La dette est aujourd'hui un outil indispensable au fonctionnement de nos économies nos économies ; c'est un peu le carburant du moteur de la croissance, mais encore faut-il que l'excès d'endettement ne vienne pas noyer le moteur ... C'est un peu ce qu'a vécu la Grèce avec une phase de réamorçage délicate et forcément poussive. Dans une entité déterminée, c'est-à-dire un pays, peut-on agréger dette publique et dette privée ou des fractions de ces deux dettes ? C'est ce que semble avancer Jean Tirole, prix Nobel d'économie, lorsqu'il déclare que la dette publique et la dette privée financière doivent être considérées comme un tout : pour lui, la dette bancaire est en réalité de la dette publique. Néanmoins, on ne peut pas aller jusqu'à soutenir la thèse des vases communicants entre dette publique et dette privée. En ce qui concerne la dette privée, chaque pays a des comportements d'épargne et d'endettement spécifiques. La situation française ne semble pas,

de la dette publique incombant à l'État- 80 % du total -six années de recettes budgétaires. Au regard de cette situation, il convient de poursuivre une politique rigoureuse de réduction des déficits et de l'endettement. C'est l'objectif que s'est fixé le Gouvernement, avec une stabilisation de la dette à 98 % du PIB en 2018 et en 2019 et une diminution vers les 90 % en 2021-2022.

oui, la dette est un instrument économique utile, et même très nécessaire. C'est vrai de la dette publique comme de la dette privée. On peut être en déficit dans une période de crise pour relancer la machine économique et protéger les plus faibles, en permettant, par exemple, au système de l'assurance chômage de continuer à fonctionner, tout comme une entreprise peut emprunter pour investir et se développer dans une phase de croissance. Cependant, on ne peut se satisfaire d'un recours systématique à la dette, quelle que soit la situation économique : pour pouvoir s'endetter en période de crise, il faut se redonner des marges quand la conjoncture est plus favorable. Tout est question de dynamique : c'est le battement entre ces périodes d'endettement et de désendettement qui permet d'avoir un modèle soutenable. Sans caricature ni confusion, portons d'abord un regard sur la dette publique. Je commencerai

ans, la France n'a jamais mis à profit les périodes de croissance pour réduire son ratio de dette. Cette tendance française fait figure d'exception dans le paysage européen. Nous sommes le seul pays de la zone euro dont le ratio de dette ne diminue pas depuis 2015, alors que l'on observe une baisse moyenne de 7 % ailleurs en Europe. Le problème vient de plus loin : voilà dix ans, nous avions le même niveau de dette que l'Allemagne ; depuis 2007, il y a divergence. L'Allemagne a réduit son ratio de dette, signe que la dette n'est pas une fatalité, tandis que la France a laissé sa dette s'envoler. Nous ne savons pas renverser la vapeur quand notre économie va mieux : ce n'est pas soutenable. La dette doit rester un outil, et non être une drogue l'addiction à la dette est un poison lent, qui risque de nous placer dans une position délicate si nous ne faisons rien. On ne marche pas sur la dette, c'est elle qui vous marche dessus si elle n'est pas maîtrisée. Il est essentiel de réduire la dette par beau temps

Depuis plus d'un an, nous avons inversé la tendance et affirmons des objectifs ambitieux. Nous avons endigué la hausse constante de la dette publique grâce à nos efforts budgétaires. Notre cap pour le quinquennat est clair : cinq points de dette en moins et un déficit public proche de zéro en 2022. Cette réduction de la dette et du déficit passe par un effort sur la dépense publique, en ciblant les postes sur lesquels des économies sont possibles, mais surtout en repensant les missions et l'organisation de l'État.

Il faut attaquer les problèmes sociaux à la racine, plutôt que de traiter leurs symptômes infinis. C'est tout le sens du travail que le Gouvernement mène actuellement sur l'éducation ou sur la formation. Il faut proposer un nouveau modèle économique avec moins de dépense publique et de dette, moins de prélèvements obligatoires, mais plus de soutien à l'investissement et à l'innovation, plutôt que de recourir sans cesse à plus de dépense publique, comme nous le faisons depuis des décennies.

La lutte contre la dette tient aussi à notre capacité à faire payer leur juste part d'impôt aux entreprises qui dégagent le plus de valeur, notamment grâce à nos données. La journée d'hier aura été essentielle dans ce combat.

Sur le long terme, nous devons aussi développer le financement en fonds propres de nos PME. C'est tout le sens des mesures du projet de loi PACTE relatives aux produits d'épargne des Français, qu'il

Mais la question de la dette n'est pas une question purement nationale. Je voudrais conclure par quelques mots sur la dimension européenne de cette problématique. Nous appartenons depuis maintenant vingt ans à une union monétaire. La monnaie commune nous a beaucoup apporté en termes de stabilité et de facilitation des échanges. Mais cette appartenance à une zone monétaire impose à chaque État membre un effort de discipline accru, car les décisions prises dans chaque capitale ont un impact sur tous. Nous prenons pleinement notre part de ces efforts que nous exigeons de tous nos partenaires. Cette zone monétaire commune doit être complétée. En effet, en l'état des choses, nous sommes mal armés collectivement pour affronter une nouvelle crise des dettes souveraines. C'est la raison pour laquelle dettes souveraines. C'est la raison pour laquelle il est urgent de finaliser les réformes de la zone euro et de renforcer la solidité du système en achevant l'union bancaire, en renforçant le mécanisme européen de stabilité, en parvenant à la création d'un véritable budget de la zone euro avec à la fois une fonction de stabilisation et une fonction de convergence. Si la dette est une nécessité économique, les crises liées à la dette n'ont rien d'une fatalité. Mais il faut faire preuve de volonté politique, au niveau national comme au niveau européen. Vous pouvez compter sur le Gouvernement pour poursuivre ses efforts dans le sillon tracé depuis maintenant dix-huit mois. Nous en avons terminé avec le débat

Débat portant sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Personne ne